Monsieur le président,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 chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Michel Berson, qui fut sénateur de l'Essonne de 2011 à 2017.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, auteur de la proposition de loi.

le 30 juillet 1953, le Congrès des États-Unis adoptait le. Il s'agissait, pour l'administration Eisenhower nouvellement installée, d'affirmer une priorité politique forte : placer les petites et moyennes entreprises au coeur du modèle de développement économique et social. Cette initiative a surtout fait de la commande publique un levier d'action stratégique, au service de la souveraineté nationale. Depuis, les États-Unis n'ont raté aucun virage technologique. Et pour cause : la loi-cadre de 1953 a déployé ses pleins effets sur le temps long. Encore aujourd'hui, l'avance américaine repose pour une large part sur la robustesse de son tissu de PME et d'ETI. en Allemagne, où l'excellence industrielle tient bien plus aux savoir-faire techniques du qu'aux performances financières des grands groupes. En France, la politique économique n'a jamais mis ce tissu d'entreprises au coeur de ses préoccupations. C'est pourquoi nous n'avons pas su développer le plan industriel, grâce à un financement à la juste hauteur, toutes les innovations que notre recherche fondamentale a su révéler sur le plan scientifique. Là se trouvent, me semble-t-il, nombre des raisons de notre décrochage. La crise sanitaire aura au moins eu le mérite de remiser- espérons-le ! -quelques idées fausses qui avaient la vie dure. Je pense ici à la lubie de la « France sans usines », répétée au cours des dernières décennies, une petite musique qui nous intimait que le pays serait plus fort dans la mondialisation s'il se privait de son appareil de production. Que de temps perdu, que d'innovations manquées, que de virages technologiques ratés à cause de cette ! Nos difficultés à produire des masques, puis notre incapacité à élaborer un vaccin nous ont définitivement convaincus du contraire. C'est heureux, d'une certaine manière, mais ce n'est pas suffisant. La nécessité de réindustrialiser notre pays fait désormais consensus. Il y va de notre souveraineté nationale, et le Gouvernement a bien pris la mesure de ces enjeux. Une part importante du plan de relance concourt d'ailleurs à cet objectif, avec notamment la baisse des impôts de production, à hauteur de 10 milliards d'euros par an. Le plan de sauvetage de l'économie, mis en oeuvre en début de crise, visait déjà la préservation de notre tissu d'entreprises. Le groupe Les Indépendants a soutenu cette approche. Sans entreprises, point de reprise ; c'était donc la bonne chose à faire. Mais, ce faisant, nous avons créé un paradoxe économique sans précédent, lequel, avec un peu de recul, apparaît flagrant. D'une part, nos finances publiques n'ont jamais été aussi dégradées qu'en 2020, avec à la fois une augmentation massive des dépenses et une diminution massive des recettes. Résultat : une hausse spectaculaire de notre endettement public de 20 points de PIB en un an à peine. D'autre part, l'épargne privée aura bondi de 200 milliards d'euros d'ici à la fin 2021. En cause : la conjonction des mesures de restrictions sanitaires et de soutien à l'économie, les premières ayant pesé sur la consommation des Français, les secondes ayant préservé leurs revenus. Autrement dit, jamais la dette publique n'a été si élevée ; jamais l'épargne privée n'a été si élevée. Face à ce paradoxe historique, nous devons éviter de percuter deux écueils.

continuer à croire que les acteurs déjà en place font très bien leur travail, et qu'il serait malvenu de remettre en question l'équilibre des choses ; espérer enfin que « la vie d'avant » finira par reprendre son cours, et que tout continuera d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le second écueil, c'est de croire que toutes les solutions aux problèmes seront incubées au 139, rue de Bercy à Paris. Nous voulons tous, au Sénat, que nos politiques économiques soient conçues à destination, mais aussi à partir de nos territoires. Mes chers collègues, j'ai cru utile d'en passer par cette longue introduction pour vous parler plus précisément de la proposition de loi que je soumets à votre examen. Ce texte n'est pas un texte de circonstances. Il est le fruit d'une longue réflexion personnelle, nourrie d'expériences professionnelles en France, aux États-Unis et en Asie, et surtout d'échanges avec les vrais faiseurs du terrain. La crise actuelle nous oblige à repenser de façon plus holistique plus holistique notre avenir économique. Face au défi climatique, les besoins d'investissement sont massifs pour accélérer la transition écologique, et le temps presse. Car l'inaction climatique coûte plus cher que la prise de mesures fortes, comme l'ont encore récemment confirmé, dans une étude parue à la fin du mois de mars, 738 économistes de l'de l'université de New York. Il nous faut redoubler d'efforts. Je vous propose donc de mobiliser l'épargne des Français vers des fonds souverains régionaux, afin de stimuler à la fois la relance économique et la transition écologique, en mode décentralisé. Le dispositif comporte deux volets : d'une part, des ressources ; d'autre part, des dépenses. Côté ressources, je vous propose d'instaurer un nouveau produit d'épargne réglementée, sur le modèle du livret A. Ce « livret de développement des territoires » doit permettre à tous les Français qui le peuvent et qui le souhaitent de savoir que leur argent contribue à financer la réindustrialisation en stimulant les écosystèmes locaux et les emplois y afférents. Côté dépenses, je propose que ces fonds souverains constituent de nouvelles ressources d'investissement à la disposition de chaque région qui en ferait la demande, sur son territoire. Le mécanisme s'appuie donc sur des savoir-faire existants : d'une part, la collecte de l'épargne par le réseau bancaire, qui pourra proposer un nouveau produit, déplafonné, et dont la rémunération dépendra de celle du livret A ; d'autre part, des élus locaux qui utiliseront la commande publique pour stimuler des écosystèmes d'innovation, faire émerger et consolider des « verticales industrielles », en développant des projets d'infrastructures et en déployant des solutions de transition écologique. Mais cette solution se fonde surtout sur une vision dynamique de la dépense publique, qui stimule le cercle vertueux croissance-emploi. Cette vision s'oppose à une lecture trop comptable, qui ne perçoit l'investissement que comme une dépense. Les débats en commission ont soulevé d'importantes questions techniques. Elles sont intéressantes et nous allons pouvoir en débattre aujourd'hui. J'en profite pour remercier M. le rapporteur pour le temps qu'il a bien voulu consacrer à l'étude de ce texte. Je regrette simplement qu'il n'ait pas fait de propositions, arguant tantôt de vices de conception technique, tantôt du si fameux article 40 de la Constitution. En tout état de cause, si j'ai compris ce que vous ne vouliez pas, monsieur le rapporteur, je n'ai toujours pas compris ce que vous vouliez Mon collègue Emmanuel Capus vous présentera tout à l'heure plusieurs amendements qui devraient répondre à certaines de vos légitimes craintes en sécurisant le dispositif et en étendant son champ d'application. Je reviendrai simplement sur le principal argument que vous avez opposé au mécanisme proposé, à savoir son présumé manque d'intérêt pour les collectivités. Les régions qui recourraient au dispositif pourraient emprunter à un taux garanti dans la limite du double du taux du livret A. Dans le contexte actuel de taux bas, le Gouvernement a fait le choix de fixer le taux du livret A au-dessus du marché, à 0,5 %. Dans le dispositif que je vous propose, les régions pourraient donc emprunter à des taux inférieurs à 1 %.

Mais souvent les taux varient, et « bien fol est qui s'y fie » ... Selon votre propre source, monsieur le rapporteur- l'Observatoire de la dette des collectivités locales -, les taux étaient en 2018 de 1,10 % et en 2014 de 2,40 %. %. Le programme de stabilité, présenté hier par le ministre Olivier Dussopt, laisse entendre que Bercy envisage peut-être une remontée des taux. En outre, la question n'est pas tant de savoir si les régions ont accès, pour financer leurs dépenses courantes, à de l'argent pas cher que que de déterminer si, pour des projets innovants d'infrastructures, les acteurs institutionnels en présence proposent des financements abordables, de la dette à taux raisonnable pour rendre économiquement viables des projets gourmands en capitaux- je pense, par exemple, aux infrastructures de transport à l'hydrogène vert.

Je veux être claire : cette proposition de loi ne vise pas à apporter une solution conjoncturelle à un problème conjoncturel ; elle vise précisément à garantir aux collectivités une solution structurelle de financement.

le meilleur temps pour réparer sa toiture, c'est lorsque le soleil brille ». Vous conviendrez avec moi, mes chers collègues, qu'il vaut mieux travailler à des solutions de financement lorsque les taux sont bas, plutôt que lorsqu'ils sont hauts.

Le premier constat tient à la forte croissance de l'épargne des Français sous l'effet des mesures de confinement. Rien que pour 2020, la Banque de France estime le surcroît d'épargne à 110 milliards d'euros, dont plus de 42 milliards sont venus gonfler l'encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire.

D'autre part, les ressources collectées sur les livrets d'épargne réglementés ne « dorment » pas, mais sont déjà mobilisées pour soutenir des politiques publiques essentielles. Le livret A, comme vous le savez, permet de financer le logement social et d'accompagner le financement des investissements publics locaux.

D'abord, l'objectif de permettre aux Français de donner du sens à leur épargne correspond à une aspiration forte de nos concitoyens, comme en témoigne le développement de nombreux labels d'investissement responsable. Ensuite, le soutien aux fonds propres des entreprises constitue le principal cheval de bataille pour les accompagner dans la sortie de crise. Nous serons d'accord sur ce point : pour les PME en particulier, un appui au niveau régional est un élément de réponse utile, et je salue à cet égard les initiatives d'ores et déjà prises par plusieurs régions en ce sens,

le fonds souverain régional envisagé s'apparente, en réalité, à un simple mécanisme d'emprunt bancaire ouvert aux régions, tandis que la lisibilité de l'utilisation de l'épargne n'est pas plus évidente que pour l'actuel livret A. Cette épargne serait collectée par le réseau bancaire, puis redistribuée sous forme de prêts, non pas en fonction des montants déposés sur ces livrets dans chacune de nos régions, mais en fonction d'une clé de répartition définie à partir du potentiel financier de chaque région.

l'article 1 crée le « livret de développement des territoires », dont les caractéristiques reprennent en partie celles du livret A : une liquidité permanente pour les épargnants, une exonération fiscale et sociale des intérêts perçus et un fléchage de la ressource. Cependant, deux différences significatives doivent être signalées : la rémunération est majorée au bout de cinq ans, tandis que la garantie de l'État n'est pas prévue. Il en résulte une majoration sensible du coût de la ressource, problématique lorsqu'il sera question d'envisager son utilisation. Ensuite, 90 % des encours collectés devraient être prêtés aux régions volontaires, en fonction d'une clé de répartition fondée sur leur potentiel financier. Le mécanisme appelle de ma part deux observations. La première concerne son coût pour les finances publiques, qualifié de « prohibitif » par le Gouvernement. Deux effets se conjuguent : une exonération ponctuelle des retraits opérés en 2022 sur d'autres produits d'épargne pour abonder le nouveau livret et une dépense fiscale majorée en raison du taux bonifié par rapport au livret A. Pour un encours de 80 milliards d'euros, cela représente tout de même une centaine de millions d'euros par an. La seconde observation concerne le fonctionnement du dispositif, qui n'est pas opérationnel en l'état. La promesse La promesse faite à l'épargnant en termes de liquidité permanente et de rémunération n'est guère compatible avec l'emploi imposé de la ressource. En dépit du fléchage de l'encours du aucune centralisation des fonds n'est prévue, ce qui aurait permis de mutualiser les risques et d'optimiser l'usage de la ressource, comme c'est le cas pour le livret A. Malheureusement, les amendements déposés ne sont pas de nature à répondre à ces difficultés structurelles.

En premier lieu, ces fonds souverains régionaux ne seraient pas dotés de la personnalité morale, ce qui les rendrait indistincts des régions du point de vue juridique et comptable. En second lieu, plutôt que d'investir dans des actifs, ils auraient surtout pour fonction de financer les dépenses d'équipement des régions lorsque celles-ci sont compatibles avec les objectifs des schémas

ensuite, et principalement, une fraction de l'encours du LDT qui serait prêtée par les banques à un taux ne pouvant excéder le double de celui du livret A. Dans la situation actuelle,

En résumé, ce ne sont pas des fonds souverains qui sont ici créés, mais bien un nouveau mécanisme d'emprunt bancaire au profit des régions afin de financer leurs dépenses d'équipement. Il n'y a là rien de très nouveau ...

Deuxièmement, compte tenu des conditions de rémunération du LDT, le taux d'emprunt servi aux régions serait proche de 1 %, alors même qu'elles s'endettent actuellement à 0,58 % en moyenne.

loi, l'un des intérêts du LDT pour l'épargnant devrait être, notamment, de pouvoir constater concrètement l'impact de son placement sur le développement régional. Ce ne serait pas possible en l'état. Si je n'ai pas été convaincu par le dispositif proposé, j'ai toutefois cherché, ma chère collègue, des pistes d'amélioration. L'une d'elles aurait été, à mon sens, de constituer de véritables fonds souverains régionaux chargés de mobiliser l'encours du LDT localement,

Concernant l'opportunité, le droit permet déjà aux régions, en partenariat avec le secteur privé et dans le respect du droit de l'Union européenne, de constituer et de doter des fonds d'investissement ou de prendre des participations directes au capital de sociétés commerciales. J'ai pu échanger avec les principaux acteurs concernés. Chaque fois, le même constat s'est imposé : le dispositif, tel qu'il est imaginé, ne fonctionne malheureusement pas et, surtout, l'objectif visé ne semble pas répondre aujourd'hui à une carence identifiée, notamment en termes d'accès des régions au crédit. En conséquence, mes chers collègues, je vous propose de rejeter cette proposition de loi.

la crise économique et sanitaire que nous traversons dessine incontestablement un paysage inédit, modifiant en profondeur les paramètres de notre économie, au premier rang desquels l'épargne des Français, qui, principalement faute de débouchés de consommation, a fait l'objet d'une importante accumulation depuis le premier confinement. Cette épargne peut être mise au service de la relance de l'économie. Nous partageons tous ce point de vue, me semble-t-il. Au cours des derniers mois, le Gouvernement a pu constater la pleine mobilisation des élus locaux et nationaux, désireux d'élaborer des solutions novatrices qui permettraient d'orienter ce supplément d'épargne vers nos entreprises pour leur permettre de rebondir plus facilement. Parallèlement, les budgets de l'État et des collectivités locales sont fortement sollicités et de nombreuses idées se font jour sur le thème d'un grand emprunt national. Pour autant, la réflexion que nous devons porter sur l'épargne doit être menée au regard du contexte macroéconomique singulier dans lequel nous nous trouvons. La crise que nous traversons n'est pas une crise financière ni même une crise bancaire : le contexte de taux d'intérêt très bas et d'offres de financement abondantes que nous connaissions avant la crise perdure, notamment grâce grâce à l'action résolue de la Banque centrale européenne. Je souhaite d'abord rappeler que les collectivités territoriales ont abordé cette crise dans une bien meilleure situation que celle qui prévalait au moment de la crise de 2008 et qu'elles bénéficient d'une offre de financement abondante, diversifiée et exceptionnellement peu onéreuse. Le taux moyen auquel les collectivités empruntent s'élevait ainsi en 2019 à 0,71 % et a continué à baisser

qui souhaitent, à juste titre, investir pour insuffler un nouveau dynamisme à leur territoire n'ont pas, à ce stade, de difficulté de financement par l'endettement qui les empêcherait d'y parvenir. Les collectivités qui veulent participer à la relance sont donc plus que bienvenues pour développer des projets d'investissement durables, en parallèle de ceux déjà menés par l'État ! Je n'ignore évidemment pas

dans son rôle de financement des territoires, répond déjà aux carences du marché privé pour financer certains besoins très ciblés. Il s'agit notamment du financement de certains projets de très long terme dans les domaines de la rénovation énergétique et des infrastructures. Au contraire, le mécanisme que cette proposition de loi instaurerait, si elle était adoptée, mettrait à la disposition des collectivités une ressource bien moins intéressante que celles qui sont aujourd'hui à leur disposition. En effet, le livret envisagé offre à l'épargnant un support parfaitement liquide et dont le capital et la rémunération sont garantis. Ces caractéristiques font de cette ressource une ressource très chère pour les collectivités et assez peu adaptée à l'investissement productif.

car on ne peut pas financer les fonds propres des entreprises avec une ressource liquide et dont le capital est garanti. Si un fonds prend des parts dans une entreprise et que celle-ci perd de la valeur, il faudra rembourser l'épargnant, et cette dépense devra être assumée par la collectivité sur ses fonds propres.

La Banque de France relève que le taux d'épargne des ménages a dépassé 18 % en 2020, alors qu'il se situait plutôt autour de 14 % les années précédentes. Une part de cette surépargne a vocation à être dépensée lorsque les possibilités de consommation seront pleinement rétablies. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que les Français ont privilégié des supports d'épargne liquide tels que les dépôts à vue ou le livret A. Ainsi, les livrets réglementés ont collecté près de trois fois plus de ressources depuis un an que l'année précédente. Toutefois,

Ce n'est pas vrai, d'une part, parce que l'épargne déposée par les Français dans les banques contribue au financement de l'économie, et donc, des collectivités et des entreprises par l'intermédiaire du crédit bancaire et, d'autre part, parce que près de 60 % des livrets A et des LDDS sont centralisés au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations qui finance déjà

s'agit du livret A. Le Gouvernement partage toutefois votre souhait, qui est juste, d'orienter encore davantage l'épargne des Français vers les territoires. Il s'est mobilisé à cette fin dans le cadre de France Relance. Bruno Le Maire a demandé à la Caisse des dépôts et consignations de faire évoluer les conditions de mobilisation de la ressource du fonds d'épargne afin d'encourager le financement du secteur public local et de la transition écologique. De plus, le lancement, le 19 octobre 2020, du label Relance a permis d'identifier les fonds d'investissement qui s'engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises, cotées ou non. les supports d'épargne grand public, chaque épargnant peut donc contribuer au soutien de la reprise économique. En contrepartie du label, les fonds labellisés s'astreignent à effectuer un reportage semestriel dans lequel ils identifient la localisation territoriale de leurs investissements dans les PME et entreprises de taille intermédiaire non cotées.

Enfin, l'action de l'État, coordonnée avec celle des régions, permettra d'apporter directement des financements en fonds propres aux entreprises. Avec l'appui de la Banque publique d'investissement, l'État abondera à hauteur de 250 millions d'euros

et être labellisés Relance. Comme vous pouvez le constater, grâce à France Relance, nous allons plus loin pour affecter efficacement l'épargne des Français au bénéfice du dynamisme économique de nos territoires, ce qui démontre que, si les moyens

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise sanitaire exacerbe les inégalités face à l'emploi, la santé ou encore au logement. Les inégalités financières sont particulièrement criantes et, de plus, elles entretiennent ces déséquilibres. Selon la Banque de France, l'épargne des Français accusait une hausse de plus de 100 milliards d'euros à la fin de 2020, et celle-ci pourrait atteindre 200 milliards à la fin de 2021, soit le double du montant du plan de relance. Il me paraît important de préciser que toutes et tous ne sont pas à égalité dans la constitution d'une telle épargne. Entre mars et août dernier, 70 % de l'épargne a été réalisée par les 20 % de ménages les plus aisés, alors que la situation des plus modestes s'est au contraire dégradée. Le Conseil d'analyse économique souligne ce double mouvement antagoniste : dans le même temps, les 10 % de ménages les plus modestes ont dû s'endetter pour assumer la diminution de leur rémunération ou, pour plus de 365 000 salariés, La proposition de loi nos collègues a le mérite de proposer la mise à disposition de nouvelles ressources pour contribuer à la relance du pays, en permettant aux Français d'en être acteurs tout en donnant des pouvoirs aux élus locaux pour orienter les investissements. Malgré tout, plusieurs interrogations nous en éloignent. La création d'un tel livret de développement des territoires serait une aubaine pour les plus fortunés qui disposent d'une épargne bien constituée et solide, et qui, de ce fait, sont en capacité de la placer à long terme et de maximiser leurs intérêts.

Si nous devons réfléchir à l'utilisation de l'épargne des Français, nous devons aussi envisager la taxation de l'épargne des plus riches sous la forme d'une imposition renforcée des tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu ou d'une contribution exceptionnelle sur la fortune et le patrimoine.

en se superposant maladroitement à l'activité de la Banque des territoires et aux ressources de la Caisse des dépôts, et cela sans centralisation. Il constitue aussi un risque pour le financement du logement social, puisque la création d'un nouveau livret pourrait favoriser une décollecte d'autres livrets qui abondent notamment ce secteur.

424 milliards d'euros : tel est le chiffre avancé avant-hier dans un quotidien national par Olivier Dussopt pour évaluer la facture globale de la crise sanitaire que nous vivons. Du sauvetage de l'économie du printemps 2020 au plan de relance qui se déploiera jusqu'en 2022, la puissance publique a mobilisé d'importants moyens financiers pour faire face à la crise du coronavirus. À l'effet de ces mesures de soutien à l'économie s'est ajouté celui de la récession sur l'encaissement des recettes fiscales. Résultat : la France a quasiment doublé en 2020 le niveau de son déficit et dégradé de près de vingt points le ratio de sa dette publique rapportée à la richesse produite. Dans le même temps, sous l'effet des mesures de restriction et des incertitudes quant à l'évolution de l'épidémie, les Français ont très fortement épargné. Forte de ce constat paradoxal et animée par le souci de mobiliser davantage de moyens dans cette crise au service de nos territoires, de nos entreprises et de leurs emplois, notre collègue Vanina Paoli-Gagin nous saisit de cette proposition de loi visant à réorienter l'épargne des Français vers l'économie dite réelle. Je partage pleinement l'idée et l'intention que sous-tend le livret de développement des territoires introduit à l'article 1 de cette proposition de loi, que j'ai d'ailleurs cosignée avec six de mes collègues du groupe Union Centriste.

D'épargne forcée au sortir du premier confinement de mars 2020, elle est devenue épargne de précaution sanctuarisée dans l'incertitude de 2021. Drainée vers l'investissement productif, elle offre une formidable possibilité de relance. La capter en intéressant les épargnants par la création de livrets attractifs, puis la mobiliser la création de fonds souverains régionaux comme le propose notre collègue permettrait d'aller plus loin dans la capacité d'investissement des collectivités locales

du groupe Les Indépendants- République et Territoires. Malheureusement, comme l'a rappelé Philippe Dallier dans son rapport, le dispositif tel qu'il est proposé ne conduit pas à créer, au sens où on l'entend habituellement, de véritables fonds souverains régionaux chargés de mobiliser l'épargne en direction du tissu économique local. Par ailleurs, d'importantes difficultés pratiques ont été mises en évidence par la commission des finances. Compte tenu des conditions de rémunération du nouveau produit d'épargne proposé, les régions se trouveraient exposées à des taux d'emprunt supérieurs à ceux qui leur sont proposés par le marché, ce qui, hélas, réduit considérablement l'intérêt du mécanisme tel qu'il a été Une piste d'amélioration fort justement relevée par notre rapporteur serait de constituer d'authentiques fonds souverains régionaux qui permettraient localement aux collectivités d'octroyer des prêts ou de prendre des participations au capital des entreprises. Cela permettrait de financer l'investissement de manière plus pertinente que ce que permettent déjà aujourd'hui plusieurs types de fonds d'investissement régionaux existants. L'obstacle principal à la faisabilité de ce dispositif, outre sa recevabilité financière par voie d'amendement, serait alors la dotation en fonds propres, nécessaire pour que ces fonds d'investissement puissent assumer leurs missions. Mais encore une fois, le ticket d'entrée s'avérerait trop élevé pour bon nombre de collectivités.

Quoi qu'il en soit, les membres du groupe Union Centriste se réjouissent aujourd'hui d'avoir l'occasion de débattre d'un dispositif, qui, bien que non abouti, soulève des réflexions qui méritent de retenir toute notre attention. Le lien entre placement financier, besoin conjoncturel de financement des collectivités et utilisation locale de la ressource doit pouvoir,

présentée par Mme Vanina Paoli-Gagin visant à orienter une partie de l'épargne des Français vers des fonds souverains régionaux met en exergue deux constats. premier est que la crise sanitaire que traverse malheureusement notre pays s'est traduite par une hausse historique du taux d'épargne des ménages, liée à la fois à la diminution des possibilités de consommation- c'est ce qu'on appelle parfois l'épargne forcée -et à la montée des incertitudes économiques qui conduit à une épargne de précaution.

la constitution d'une surépargne de 200 milliards d'euros, soit près de 8 % du PIB. Il s'agit d'une épargne de court terme, déposée sur des comptes courants et les livrets d'épargne réglementée, alors que des supports à échéance plus longue seraient plus adaptés aux besoins de financement de notre pays. En effet, les fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises constituent le meilleur moyen pour soutenir les entreprises et les accompagner dans la sortie de crise. À cet égard, un appui à l'échelon régional peut constituer

Je partage donc le souhait de créer un fonds qui puisse coordonner les interventions financières des collectivités publiques situées dans le ressort territorial de la région en lien avec tous les acteurs locaux, en particulier les collectivités territoriales, afin d'assurer le financement des investissements en faveur de la redynamisation et de l'attractivité de nos territoires, de la réindustrialisation au désenclavement des territoires ruraux, de leur adaptation au changement climatique au développement des mobilités,

En effet, les ressources collectées sur les livrets d'épargne réglementée sont déjà mobilisées pour soutenir des politiques publiques essentielles. Ainsi, comme vous le savez, le livret A finance le logement social. Dans un contexte de grande tension sur le marché du logement et de paupérisation d'une grande partie de nos concitoyens, on peut donc légitimement s'inquiéter que le LDT proposé concurrence le livret A et risque d'affecter la dynamique de production de logements sociaux. Par ailleurs, on sait que cette surépargne concerne principalement les ménages aisés. En effet, le Conseil d'analyse économique indique que les 20 % des ménages aux revenus les plus élevés ont 70 % de l'épargne supplémentaire. L'outil proposé ne répond donc pas au problème majeur de notre société qu'est l'accroissement des inégalités, creuset de la désagrégation sociale et du délitement de la promesse républicaine. Nous devons y remédier, car c'est l'un des grands enjeux actuels. socialiste a d'ailleurs récemment fait des propositions en ce sens. Pourquoi ne pas mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour cofinancer l'effort exceptionnel de l'État pour lutter contre les conséquences de l'épidémie de covid-19, en instaurant un impôt sur le capital en supprimant la taxe forfaitaire sur les dividendes ? La réponse doit être simple et directe, à savoir une taxation exceptionnelle des revenus ayant bénéficié aux foyers les plus riches et aux entreprises dont les profits ont explosé. Cela permettrait de cofinancer les mesures de soutien aux ménages, aux entreprises et aux mouvements associatifs fragilisés par cette crise et de les accompagner dans leur transition vers des pratiques plus durables. Par ailleurs, on constate dans les territoires, en particulier ruraux, un niveau d'encours de dette très nettement inférieur au montant de l'épargne des acteurs locaux. Il en résulte que, de manière paradoxale, les territoires qui ont un fort besoin d'investissement financent des territoires qui ont un fort niveau d'investissement, de développement et de moyens. Il y a donc lieu aujourd'hui, en vue de favoriser la cohésion territoriale, de mettre en place des circuits courts en matière de financement. C'est aussi cela, le développement durable. Dès lors, il pourrait être envisagé d'obliger les banques à investir sur les territoires une part importante des sommes collectées sur ces mêmes territoires. Nous pourrions à cet égard nous inspirer de la loi sur le financement communautaire, qui est un dispositif législatif américain américain portant sur les relations entre les banques et d'autres grands organismes financiers et les territoires. Cette loi revêt par certains aspects un caractère unique dans la mesure où elle contraint les banques à rendre compte de la politique qu'elles mènent sur les territoires et les incite à prêter aux habitants et aux entreprises les plus fragiles. Elle nous apporte un éclairage sur le potentiel que constitue l'engagement volontariste des banques pour le développement économique et social des territoires en panne de croissance. ans, le dispositif a mobilisé plus de 1 400 milliards de dollars de crédits et de services bancaires au bénéfice de territoires et de populations fragiles pour promouvoir le développement local

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à la mi-février, notre commission des finances débattait de la mobilisation de l'épargne en faveur de l'économie. Début mars, Bruno Le Maire indiquait que le Gouvernement travaillait à des incitations qui permettraient aux Français de dépenser leur épargne dans l'économie, et donc de participer à la relance économique. Fin mars, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes annonçait le lancement d'un fonds souverain régional pour investir dans des entreprises qui pourraient même collecter l'épargne des Français sous réserve d'un agrément par Parlementaires, ministres et élus locaux s'accordent sur la nécessité de mobiliser l'épargne des Français en faveur de la relance. C'est un consensus politique frappé au coin du bon sens. Ce matin,

C'est pourquoi ce dispositif, qui est structurel et non conjoncturel, peut parfaitement s'avérer utile. Le deuxième problème

troisième problème est la liquidité du livret. On nous indique qu'on ne finance pas des prêts à long terme avec une épargne liquide. Très bien.

Soit. Soyons très clairs : l'objectif de ce texte n'est pas de remettre en question le financement du logement social. Il est de permettre aux Français qui le veulent et qui le peuvent de participer au financement de la relance autrement qu'en créant de la dette qu'ils finiront par payer de leur impôt, et de le financer au plus proche de chez eux sur leur territoire. C'est

chers collègues, en présentant cette proposition de loi, nous avons pris la responsabilité de proposer une solution concrète plutôt que d'ouvrir un simple débat. Nous faisons confiance au débat parlementaire pour muscler le dispositif. J'espère que vous y participerez.

la crise sanitaire met à mal notre idéal d'égalité. Cela se reflète tout particulièrement dans la répartition de l'épargne dont il est question dans cette proposition de loi. Une partie de la population dont la vie professionnelle ne tenait qu'à un fil a subi de plein fouet et sans filtre les conséquences économiques du confinement : les petits indépendants et autoentrepreneurs, les intermittents de l'emploi et les chômeurs déjà privés d'emploi avant la crise. De l'autre côté, les stables, les détenteurs de capitaux économiques qui ont la chance d'être bien installés ont largement surépargné et constitué par la même occasion un patrimoine financier supplémentaire. D'après une étude du Conseil d'analyse économique qui a déjà été largement citée, 20 % des 20 % des ménages aux revenus les plus faibles ont vu leur épargne diminuer, alors que la moitié du surcroît d'épargne a été réalisée par 10 % des ménages les plus aisés.

Si nous notons avec intérêt l'envie de préparer l'avenir, y compris en termes de transition écologique, il nous semble que des garanties devraient être apportées pour que ces crédits soient fléchés vers l'économie sociale et solidaire, sujet qui intéressera sans doute

Les deux axes qui servent d'architecture à la proposition de loi ont le mérite d'être intéressants. Il s'agit, d'une part, de créer un nouveau livret d'épargne, d'autre part, d'utiliser la ressource collectée par les régions. du nouveau livret d'épargne, la proposition de loi suggère la création d'un livret de développement des territoires qui permettrait de financer des fonds souverains. Celui-ci concurrencerait donc le livret A

bien observer ces quelques éléments, chacun peut présager que le livret de développement des territoires sera beaucoup plus attractif que le livret A. Or cette attractivité risque de diminuer fortement les encours sur le livret A, alors qu'ils servent

d'équipement. Or les régions n'ont pas de difficulté pour accéder au crédit. Rappelons aussi que le droit en vigueur permet déjà aux régions de doter des fonds d'investissement. Des dispositifs existent, dans lesquels les régions interviennent dans un cadre précis, avec des partenaires privés et selon des règles fixées par le droit de l'Union européenne. Enfin, les régions peuvent déjà prendre des participations au sein des sociétés commerciales et accorder des prêts ou des avances remboursables. Votre amendement n° 5 rectifié, madame Paoli-Gagin, vise à ouvrir aux fonds souverains régionaux la possibilité d'investir en fonds propres

Ils ajoutent une nouvelle strate administrative chargée de piloter les investissements publics sans justifier réellement son existence. Autrement dit, ils complexifient l'organisation des régions sans renforcer leur capacité réelle d'investissement.

la bonne utilisation de l'épargne constituée par les Français depuis un an de restrictions liées à la pandémie est un vrai défi. La proposition de loi présentée par notre collègue Vanina Paoli-Gagin tente légitimement d'y répondre. En dehors dehors de ce contexte exceptionnel, l'orientation de l'épargne par le marché ou par la puissance publique est toujours un objet de débat. En témoigne le cas de l'assurance vie,

Par ailleurs, les épargnants sont souvent soucieux de donner du sens à leurs placements, au-delà d'objectifs de pure sécurité ou de rentabilité financière. Les particuliers se voient ainsi proposer des produits dotés de labels d'investissement responsable ou de développement durable. Les restrictions liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 ont fortement fait chuter la consommation des ménages depuis un an, ce qui a entraîné, pour un certain nombre d'entre eux, une surépargne. Estimée entre 100 milliards et 120 milliards d'euros en 2020, en 2020, celle-ci pourrait atteindre 200 milliards d'euros à la fin de 2021. La question se pose donc de trouver les meilleurs moyens de placer et d'utiliser cette épargne supplémentaire. Je citerai, à titre d'exemple, la proposition de loi déposée l'an dernier par mon collègue Éric Gold, qui prévoyait l'institution d'un grand emprunt national de 50 milliards d'euros pour le financement du système de santé et des autres politiques publiques. Cet emprunt aurait été ouvert à la souscription des particuliers. La proposition de loi que nous examinons tend à créer un nouvel instrument de financement des politiques régionales, par le biais de fonds souverains régionaux, qui seraient principalement financés par la collecte d'un nouveau produit d'épargne appelé « livret de développement des territoires Ces nouvelles lignes budgétaires serviraient, en particulier, à financer des projets d'infrastructures et à mettre en place un plan de relance décentralisé, complément territorial de l'actuel plan de relance gouvernemental voté en loi de finances. La commission des finances, qui a examiné le texte il y a deux semaines, s'est montrée particulièrement sévère. En effet, si le dispositif mérite sans doute d'être amélioré, il convient néanmoins de saluer cette initiative, alors qu'il est nécessaire de mobiliser les énergies et les bonnes volontés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, dont nous ne sommes pas encore sortis- faut-il le rappeler ? Très bien ! Le nouveau livret de développement territorial aura pour principale caractéristique d'offrir une rémunération de plus en plus intéressante au fil du temps, afin d'inciter les particuliers à y placer leur épargne dans une logique de long terme. J'ai néanmoins déposé un amendement visant à préserver l'encours du livret A, qui sert à financer le logement social et le renouvellement urbain dans notre pays. effet, d'éviter un risque d'éviction vers le livret de développement territorial. Ne pourraient ainsi être retirées d'un livret A que les sommes excédant la moitié du plafond de ce dernier. Il me semble que cette condition est importante pour mettre en place le LDT sans fragiliser le livret A.

En conclusion, compte tenu de ces différentes remarques, les membres du RDSE se partageront entre un vote favorable et quelques abstentions. La parole

un prêt rebond, un fonds d'investissement « Normandie Rebond », une aide aux entreprises qui ont contracté un prêt garanti par l'État (PGE), un fonds régional de garantie, mais aussi de l'investissement direct pour soutenir le tissu économique local.

Forts de ce constat, les auteurs de la proposition de loi ambitionnent de mobiliser cette épargne des fonds souverains régionaux, dont l'objet serait d'investir dans la modernisation des infrastructures des territoires, afin d'accélérer la transition écologique et le développement économique. Posons-nous les bonnes questions : quel est le besoin des entreprises et comment le satisfaire ? À la fin de cette crise sanitaire, la trésorerie des entreprises sera, ou aura été utilisée pour éponger la dette covid. Les PME et les ETI n'auront plus de trésorerie pour investir et relancer l'économie, alors qu'il s'agit bien là d'entreprises régionales. Il est à noter que, depuis le début de la crise, 30 % des ETI ont déjà été approchées par des fonds spéculatifs. Il est urgent de renforcer leurs fonds propres pour les préparer à la reprise. Le choix a été fait, d'une part, d'encourager la relance de la consommation des ménages, d'autre part, de relancer l'investissement en entreprise les prêts participatifs et l'actionnariat des salariés,

Cependant, la difficulté à mobiliser cette épargne de précaution est liée au rétablissement de la confiance. Les Français craignent pour leur emploi, leur santé et leur retraite. Il faut donc leur proposer un placement garanti, très liquide, peu taxé, et qui offre une rémunération supérieure à l'épargne classique.

L'autorisation accordée par l'AMF permettra d'y inclure le recours à l'épargne publique locale. Concernant la proposition de loi que nous examinons, outre son coût élevé pour les finances publiques et les doutes quant à son caractère opérationnel, le modèle proposé n'a pas pour vocation de renforcer

Attendons donc les premiers retours des régions qui ont mis en place des fonds souverains régionaux, sur le modèle de ce qui existe déjà dans d'autres régions européennes. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains ne votera pas ce texte. La

vise à créer des fonds souverains régionaux, afin d'orienter l'épargne des Français vers des projets locaux. En effet, une hausse record de cette épargne a été enregistrée ces derniers mois, en raison de la crise sanitaire. L'intention est louable, et le dispositif proposé semble à première vue séduisant. En tant que conseiller régional, j'ai forcément été intéressé par des mesures dont l'objet est d'offrir de nouvelles possibilités de financement aux régions, d'autant plus qu'elles permettraient de faire participer les Français à la relance, et de financer des projets locaux. en détail le dispositif et la manière dont les régions financent leurs projets, il apparaît que le mécanisme présente des lacunes qui ne me semblent pas pouvoir être rattrapées, et que le besoin de financement des régions est à relativiser.

que les régions sont intéressées par des dispositifs d'épargne territorialisés ainsi que par le fléchage des ressources disponibles vers les fonds propres des entreprises, le livret de développement des territoires ne permet en réalité ni l'un ni l'autre. D'une part, le LDT est réparti au niveau national selon une clé liée au potentiel financier des régions. Il n'y a donc pas réellement de territorialisation. D'autre part, le fonds a principalement vocation à financer des dépenses d'équipement, pour lesquelles les régions n'ont pas de mal à trouver des financements. Le besoin que

cette lacune. Le texte ne permet pas non plus d'offrir aux régions des moyens de financement plus intéressants que ceux dont elles disposent déjà. En effet, les régions s'endettent à un taux d'intérêt évalué, en moyenne, à 0,58 %. Or les conditions de rémunération du LDT conduiraient les banques à proposer des taux d'environ 1 %, et donc moins intéressants. régions ne constatent pas plus que les établissements bancaires de carences d'accès à des financements, qui auraient pu justifier qu'elles s'endettent à des taux plus élevés. Enfin, le dispositif aurait des effets négatifs non seulement sur les finances publiques, en raison des risques d'optimisation fiscale et de la possibilité de cumuler les LDT, mais aussi sur les finances régionales, puisque le volume du prêt consenti aux régions ne serait pas négociable, ce qui pourrait conduire celles-ci à s'endetter plus que de besoin. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas favorable à l'adoption de ce texte. En revanche, il me semble qu'il serait opportun d'effectuer un bilan des moyens dont les régions disposent pour participer au capital d'entreprises. En identifiant leurs lacunes, on pourrait ensuite proposer des améliorations. L'examen de cette proposition de loi aura eu le mérite d'attirer notre attention sur un sujet important, et de nous permettre d'engager une réflexion sur la manière dont nous pourrions renforcer les dispositifs existants. La discussion les dispositifs existants. La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

En effet, compte tenu du taux actuellement pratiqué pour ce dernier, à hauteur de 0,5 % depuis le 1 février 2021, de ceux envisagés pour le nouveau livret de développement des territoires, ainsi que des facilités fiscales de retrait des fonds, il existe un risque d'éviction de l'épargne du livret A vers le livret de développement des territoires.

constitutionnel, parce que l'on réserverait ce livret de développement territorial, au taux plus rémunérateur que le livret A, à une catégorie de Français, et que l'on en exclurait une autre.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à répondre à une partie des critiques émises par M. le rapporteur, quant à la stabilité financière du dispositif proposé.

Le dispositif prévoit, toutefois, un mécanisme de sécurité qui limite ce risque, en permettant aux banques de conserver jusqu'à 10 % de l'encours déposé sur le livret de développement des territoires. Cet amendement a pour de porter ce « matelas de sécurité » à 20 %, en vue de renforcer cette protection.

les régions et les autres collectivités territoriales empruntent sur quinze ou vingt ans, et parfois sur des durées plus longues, en fonction des investissements qu'elles ont à réaliser. Le fait de ramener de 90 % à 80 % la part réservée à ce fonds souverain régional,

à la région, mais aussi à toutes les collectivités territoriales et intercommunalités.

Par ailleurs, sur le plan technique, comme l'a dit le rapporteur, un tel mécanisme devrait être organisé afin que les droits de tirage donnés à l'ensemble des collectivités locales soient bien coordonnés. Cette organisation reviendrait, en réalité, à recréer en quelque sorte une banque des territoires qui organiserait et instruirait les prêts consentis à chacune des collectivités territoriales. Or la banque des territoires existe déjà. Elle assure les besoins de financement des collectivités qui ne sont pas couverts par les financements bancaires de marché. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement

monsieur le rapporteur,

Je vous remercie